de restaurer un haut niveau de production et de réhabilitation des logements HLM. Or, il y a urgence ! En outre, le dispositif doit être revu fin 2022

Initialement prévue pour une somme de 1,5 milliard d'euros annuels, celle-ci sera réduite les premières années grâce à l'intervention du Sénat et à la mobilisation des acteurs du logement social et des associations nationales d'élus.

Et ce n'est pas rien, car le montant de la RLS équivaut chaque année à 4,5 % des loyers versés ! Qui plus est, la Cour des comptes explique que les organismes qui accueillent le plus d'allocataires APL et qui pratiquent les loyers les moins élevés sont les plus touchés. La RLS étant forfaitaire, plus les loyers sont faibles, plus son incidence est forte. En clair, plus le logement est social, plus il paie. Nous l'avions souligné tous ensemble, ici même, dès la loi de finances pour 2018, et la pseudo-mutualisation promise n'y a rien changé. Oui, la RLS a eu des effets négatifs sur le niveau de la construction, des réhabilitations et des loyers de sortie. La chute de la construction a commencé en 2018, année de sa mise en place, et donc avant la crise du covid. Elle se confirme depuis. Les municipales et le coronavirus ont bon dos ! Au-delà des chiffres, la Cour des comptes observe que la perte

Cour ajoute que les dépenses d'entretien courant, en particulier de gros entretien, ont diminué de 7 % en valeur et que, si cette baisse devait perdurer, elle provoquerait une détérioration des bâtiments et une perte d'attractivité du logement social. Déjà, dans de précédents rapports, la Cour avait insisté sur l'importance de cet entretien, en particulier de la politique de la ville. Le Gouvernement ne peut pas faire l'autruche sur ces réalités. À elles seules, elles justifieraient l'abandon immédiat de la RLS pour relancer une production soutenue de logements sociaux avec des niveaux de loyers plus bas et pour assurer un entretien et des réhabilitations réguliers La RLS menace l'avenir du mouvement HLM et de ses finances. Dès sa création, nos rapporteurs prévoyaient une détérioration de la situation financière des organismes de logement social (OLS) faisant peser de lourdes menaces sur l'avenir. La Cour constate que l'incidence financière a pu être amortie jusqu'à présent- j'y reviendrai -, mais que la RLS diminue mécaniquement les résultats des organismes. Si le potentiel financier des bailleurs reste quasiment stable, l'autofinancement du secteur HLM a néanmoins diminué, conduisant à une réduction des investissements. Elle s'inquiète pour l'avenir et estime qu'il importe d'évaluer l'impact global de la RLS sur le modèle économique et financier des HLM,

Il faut ajouter que, du fait du désengagement de l'État dans les aides à la pierre, les fonds propres sollicités pour les opérations sont passés de 5 % à 15 % entre 2000 et 2018. C'est l'asphyxie des organismes HLM qui est ainsi programmée avec la RLS.

Nous avions déjà souligné les graves conséquences de ce transfert, de fait, d'une dette de l'État vers les organismes HLM. Si ce mécanisme ne change en rien l'endettement réel de la France,

banaliser et de financiariser le logement social, comme certains gouvernements libéraux, dans d'autres pays, l'ont fait voilà des dizaines d'années. Les mêmes, aujourd'hui, font marche arrière

différentes mesures de « compensation » ne sont en rien durables, alors que Bercy et le Gouvernement souhaitent pérenniser, voire sans doute accroître la RLS. Mes chers collègues, nous devons nous y opposer et demander l'abandon de la RLS

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, pendant dix-sept ans, j'ai eu le plaisir de présider le premier bailleur social du département du Gard, comprenant 16 000 logements, dont la moitié se situe en quartier prioritaire. La question de la mixité sociale au sein de ces quartiers, où l'on comptabilise plus de 40 % de demandeurs d'emploi, représente un enjeu important. Si la nécessité de produire plus de logements sociaux semble une évidence pour beaucoup, de nombreuses contraintes demeurent

Depuis la loi de finances pour 2018, la création de la RLS vient très nettement amputer leurs recettes, et les mécanismes de compensation mis en place depuis lors sont loin d'être suffisants, Les prix du foncier sont élevés, les coûts de construction augmentent et la RLS vient alourdir l'addition. C'est notre capacité à produire de nouveaux logements sociaux qui est remise en cause. Les bailleurs les plus solides financièrement peuvent encore faire face, mais, de jour en jour, ils épuisent leurs trésoreries et leurs fonds propres. Cette situation ne pourra pas perdurer. Nous devons répondre à la demande et produire plus de logements sociaux. Pour autant, cette priorité ne doit pas nous faire oublier ou négliger nos locataires actuels. Le parc HLM existant est aujourd'hui dégradé. Les constructions des années 1970 ne correspondent plus aux conditions de vie actuelles la mixité sociale n'est plus présente ; le parcours résidentiel n'existe plus ... L'entretien et la rénovation de notre parc représentent donc un enjeu majeur. Depuis 2005, j'ai pu participer aux opérations de rénovation urbaine dans mon département

Il est urgent, madame la ministre, d'apporter des réponses politiques pour ne pas laisser prospérer un sentiment d'abandon chez les locataires du parc actuel. Pour changer l'image du logement social, nous devons commencer par changer celle de notre parc existant C'est un sujet décisif, car nos politiques en la matière peuvent avoir des répercussions positives dans de nombreux domaines. En portant une ambition pour le logement social, on agit directement sur la qualité de vie des Français, mais aussi sur leur pouvoir d'achat. Habiter un logement social, c'est économiser en moyenne 250 euros par mois de loyer. Agir sur le logement social, c'est aussi oeuvrer pour la transition énergétique que notre pays doit engager. On peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre et faire baisser la facture énergétique des ménages les plus modestes. Là encore, un signal pourrait être envoyé en rendant les bailleurs sociaux éligibles à l'ensemble des crédits d'État liés aux rénovations thermiques. Enfin, alors que la crise sanitaire a eu de sévères répercussions sur l'activité de nos entreprises, la question de la relance économique est au coeur de nos préoccupations. Une réelle ambition et un véritable plan d'investissement en matière de logement social contribueraient à redynamiser l'économie et favoriseraient l'emploi. toutes ces raisons, nous devons saisir l'opportunité de faire du logement social une politique publique prioritaire et nous donner les moyens d'atteindre nos objectifs.

De surcroît, la législation récente favorise la constitution d'entités plus importantes. Je pense notamment à la constitution des sociétés de coordination Madame la ministre, à l'heure où la crise sanitaire tend à renforcer les inégalités, il est urgent de s'interroger sur la RLS et sur les choix politiques qui ont été faits ces dernières années. La

à présent ? Trois ans après la décision du Président de la République de réduire de 5 euros les aides personnalisées au logement et d'imposer une réduction des loyers aux bailleurs sociaux, les résultats sont là : moins de 90 000 logements sociaux ont été agréés en 2020, contre plus de 120 000 en 2016. Le virus, les élections municipales et les maires réfractaires ont bon dos. En réalité, c'est bien à la suite des décisions de 2017 que la courbe s'est infléchie et c'est bien la politique du Gouvernement qui en est la principale cause. une ponction de 1,3 milliard d'euros, a considérablement affaibli les capacités des bailleurs sociaux, aussi bien pour entretenir leur patrimoine que pour investir dans de nouveaux logements. Ces mauvais chiffres ne sont pas conjoncturels, ils sont bien le résultat d'une stratégie délibérée du Gouvernement. Le logement a été identifié en 2017 comme une source d'économies pour rétablir l'équilibre des finances publiques. C'est un fait.

Selon le rapport annuel du compte du logement, publié fin 2020, les aides au logement sont passées de 2,2 % du PIB en 2010 à 1,6 en 2019. Si le logement en a été la cible privilégiée, c'est parce qu'on a estimé, au sein de l'État, que la France dépensait trop et mal pour le logement et qu'il fallait changer de modèle. Les restrictions budgétaires décidées sont un puissant aiguillon pour constituer de grands groupes de bailleurs sociaux, qui pourront ainsi ouvrir leur capital et se financer sur les marchés. Cela rend possible la remise en cause des ressources dédiées au secteur. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous constatons à travers les attaques contre Action Logement et la participation des entreprises à l'effort de construction ? Par ailleurs, les économies réalisées sur les APL diminuent leur caractère solvabilisateur et constituent une étape vers leur forfaitisation et leur dilution dans un futur revenu universel. L'erreur stratégique étant commise, comment peut-on la réparer ? Certaines solutions ont déjà été mises en oeuvre par le Gouvernement, et je lui en donne acte. Quelque 500 millions d'euros

pour la construction de 250 000 logements sociaux d'ici à 2022, Action Logement mobilisera près de 1 milliard d'euros dans le cadre de son plan d'investissement volontaire, tandis que la Banque des territoires portera son enveloppe de titres participatifs de 700 millions à 1 1 milliard d'euros. Toutefois, au moment où doivent débuter des négociations pour l'après-2022, on ne peut se satisfaire de la reconduction de l'existant, à l'exception technique de la situation des bénéficiaires de la RLS qui ne touchent pas les APL. Comme le recommande la Cour des comptes, il faut réaliser un véritable audit de la viabilité à long terme des bailleurs sociaux. Pour ma part, je pense qu'il faut aller au-delà et explorer au moins trois pistes supplémentaires.

Deuxièmement, il convient de protéger le logement social des effets de l'objectif « zéro artificialisation nette », qui va renchérir le coût du foncier. Faut-il créer une exception pour le logement social ? Ne serait-il pas temps de réexaminer le zonage qui régit les subventions des opérations et qui n'a pas été revu depuis 1978 ? nous devons encourager les maires bâtisseurs, qui sont aujourd'hui pris en tenailles entre les exonérations d'impôts locaux et les coûts d'accueil de logements sociaux. foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les nouvelles constructions sont très attendues, madame la ministre. Au total, c'est un véritable changement de cap que nous demandons, afin d'assurer, face aux défis du XXI siècle, la viabilité du modèle français de logement social, social, conçu après-guerre pour offrir un logement abordable et décent au plus grand nombre de Français, et pas seulement aux plus démunis.

Cette mesure, adoptée dès la loi de finances pour 2018, consiste en une remise de loyer financée par les bailleurs sociaux. Son principal objectif est de réduire le coût des APL pour l'État. Il est aujourd'hui nécessaire d'ouvrir le débat sur cette mesure, et ce pour au moins deux raisons. La première, c'est le recul dont nous disposons aujourd'hui pour évaluer cette mesure.

Sur ce premier point, le référé rendu public par la Cour des comptes début mars apporte de précieux éclairages. Si la Cour constate que des économies ont été réalisées pour le budget de l'État, notamment en 2018 et 2019, elle remarque également que ces économies ont été moins importantes que les objectifs initiaux, puisqu'elles se situent entre 800 et 900 millions d'euros par an, contre 1,5 milliard d'euros initialement prévus. De surcroît, elle explique que si ces économies ont été bénéfiques pour le budget de l'État, elles ont néanmoins eu des effets très négatifs pour les bailleurs sociaux, qui ont subi des pertes de ressources préoccupantes.

Le Gouvernement a annoncé la stabilisation de la RLS jusqu'en 2022, mais force est de constater que cela ne suffira sans doute pas pour relancer le logement et les investissements, 2020 a été une année noire pour le logement social. Un triste record a été atteint, seuls 90 000 logements ayant été agréés au cours de l'année. On a même constaté un recul d'activité à deux chiffres dans certaines régions, notamment en zones tendues. Compte tenu de ces deux éléments- évaluation de la mesure et crise économique -, il paraît légitime de remettre en question la pertinence

il faut aussi mettre en place des outils d'analyse partagés pour mesurer ses effets réels sur la situation financière et sur les capacités d'investissement des bailleurs sociaux. Je voudrais, en guise de conclusion, contribuer à la réflexion sur ces outils d'analyse. Les acteurs de terrain sont nombreux à nous indiquer que la RLS a été une fausse bonne idée.

à quitter les logements sociaux, notamment en dehors des zones tendues et en milieu périurbain et rural. Le logement social manque à sa vocation initiale s'il ne favorise pas la mixité sociale. Je pense que nous nous efforçons tous dans cet hémicycle de défendre cette mixité. Notre groupe souhaite donc la révision de la RLS pour maintenir la capacité d'investissement des bailleurs sociaux.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le groupe CRCE et l'ancienne ministre Marie-Noëlle Lienemann de nous proposer ce débat sur la RLS, un

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je tiens à réaffirmer tout mon attachement au modèle français du logement social et à souligner l'importance de l'action de ceux qui, tous les jours, mettent en oeuvre la politique sociale du logement. Cette politique incarne la volonté de donner un logement digne à celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'en trouver un sur le marché privé. Cette action est d'autant plus déterminante qu'elle conditionne l'efficacité d'un bon nombre de politiques publiques, qu'il s'agisse de l'accès à l'emploi, de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion ou encore de la santé. Aussi est-il important de préserver le modèle français du logement social. Toutefois, le préserver ne signifie pas que nous devrions être réduits à l'immobilisme, puisque la problématique du logement est elle-même dynamique. En effet, les besoins en termes de logements sont fluctuants. Ils varient selon des exigences sociétales en constante évolution. L'offre de logement social doit donc pouvoir, elle aussi, se réinventer et s'adapter. Le logement social a dû ainsi intégrer l'enjeu environnemental. Il compte d'ailleurs aujourd'hui parmi les secteurs stratégiques de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Il doit également faire face aux effets du vieillissement de la population. Pour répondre à ce défi de l'âge, c'est tout l'habitat social qui doit être conçu de manière plus inclusive. Il s'agit aussi de répondre à un besoin appelé à perdurer. C'est ce qui nous amènera prochainement à réfléchir à la pérennisation des objectifs de la loi SRU au-delà de 2025. Ainsi, préserver le modèle français du logement social ne signifie pas que celui-ci doive rester figé. Bien au contraire ! Le préserver, on l'a vu, c'est être capable de le faire évoluer, de l'adapter aux exigences de son époque. Le préserver, c'est aussi être capable de le moderniser de manière à le rendre plus efficace. C'est dans cet esprit qu'a été envisagée en 2018 la réduction de loyer de solidarité, réponse d'ailleurs aux recommandations de plusieurs rapports de la Cour des comptes qui appelait à une rationalisation de la dépense publique en matière d'aide au logement. La RLS consiste, je le rappelle, en une remise de loyer pour les locataires éligibles, sous condition de ressources. À cette réduction de loyer correspond une baisse quasi équivalente du montant des APL versées aux locataires concernés. Cette réduction étant financée par les bailleurs sociaux, elle a permis- et elle permet encore -à l'État de réduire la charge que représente le coût des APL pour les finances publiques. La question sous-jacente à notre débat est donc celle de l'avenir de notre modèle de logement social. Celui-ci est-il véritablement menacé par la RLS, qui pèse entièrement, c'est vrai, sur les bailleurs sociaux ? Si la Cour des comptes, dans son référé du mois de décembre, juge sévèrement ce dispositif, elle reconnaît dans le même temps que la RLS « a permis une nette réduction des dépenses de l'État pour le financement des APL, concourant ainsi au respect de la trajectoire budgétaire de la France Près de trois ans après l'entrée en vigueur du dispositif, force est de constater que le secteur a bien été en mesure d'absorber la réforme. À quel coût ! En effet, les bailleurs sociaux ont su mettre en oeuvre une gestion plus active et plus efficace de leur parc et générer les économies budgétaires attendues, sans que cela nuise aux allocataires, qui en ont même profité. J'ajoute que le secteur a bénéficié de mesures d'accompagnement, comme le gel du taux du livret A et la baisse du taux de TVA à 5,5 % pour les prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) et les opérations liées au nouveau programme national de renouvellement urbain. Il a aussi bénéficié du soutien de la Banque des territoires. Toutefois, si les bailleurs sociaux se sont révélés en capacité, avec le soutien de l'État, d'absorber la charge que représente la RLS, rendu possible en grande partie par l'état des comptes du secteur, qui présentaient alors une grande capacité d'autofinancement. C'est notamment sur celle-ci qu'a entièrement reposé l'amortissement de la première année de RLS, près de 800 millions d'euros. Aussi peut-on légitimement s'interroger sur la soutenabilité à long terme de ce dispositif, ainsi que sur la nécessité d'y apporter des modifications. Autrement dit,

une dénomination pour le moins paradoxale, dès lors que ce dispositif consiste à faire supporter aux bailleurs sociaux une partie du budget des APL. En fait de solidarité, il s'agit donc, ni plus ni moins, d'un mécanisme de transfert de charges de l'État vers le secteur du logement social. Vouloir porter atteinte à une aide en faveur des personnes en difficulté, quand bien même l'atteinte serait modique et compensée, pose question dans son principe même : cela fait peser un regard culpabilisant sur les personnes qui en bénéficient et plus généralement sur notre système de solidarité, trop souvent pointé du doigt comme excessivement coûteux. C'est là un parti pris regrettable et une perte d'énergie. Or cette énergie serait sans doute mieux employée à trouver des solutions efficaces et adaptées pour remédier à la précarité qui s'est durablement installée dans notre pays.

des économies substantielles, le procédé n'en est pas moins insidieux, puisqu'il salue la réalisation d'un second objectif : inciter les organismes HLM à une gestion plus efficace de leur parc. En clair, le ministre semble nous dire que les bailleurs n'étaient ni efficaces ni économes.

auraient permis des investissements de l'ordre de 50 à 70 millions d'euros en faveur de la réhabilitation, en particulier thermique, ou de la construction neuve. Pour se projeter, les bailleurs doivent pouvoir s'appuyer sur une politique de loyers stable et prévisible. Or, avec l'introduction de la réduction de loyer de solidarité, le Gouvernement a instillé l'aléa réglementaire et la crainte d'une baisse arbitraire et unilatérale des loyers dans un contexte où le secteur avait déjà dû absorber des mesures d'ordre budgétaire, comme sa contribution à la Caisse de garantie du logement locatif social,

L'État a d'ailleurs concédé son erreur, puisque, dans le cadre des concertations menées avec les représentants des bailleurs, il a accepté de renforcer les mesures de correction et de compensation, alors que, dans le même temps, Action Logement proposait un plan d'investissement volontaire pour accompagner le secteur. Alors, n'a-t-on pas là, finalement, l'illustration de la fausse bonne idée : contestable dans ses fondements, complexe dans sa mise en oeuvre, limitée dans ses effets ? Mon propos n'est pas de défendre l'inaction ni de nier la nécessité de réaliser des économies, ici comme dans d'autres secteurs. C'est la méthode que l'on peut critiquer : pointer du doigt ; opposer les catégories entre elles consulter sans réellement concerter ni entendre ; précipiter la décision sans attendre les conclusions de l'étude d'impact préalable ; concéder des ajustements plutôt que remettre en cause. La Cour des comptes sollicite une évaluation de cette réforme. Celle-ci doit être rapide, en particulier pour appréhender les effets du nouveau mode de calcul des APL, entré en vigueur le 1 janvier de cette année et consistant à prendre en compte en temps réel l'évolution des ressources des allocataires, ce qui conduira à procéder plus fréquemment à des ajustements de la RLS. Surtout, la construction de cette évaluation doit se faire avec la bonne méthode : il faut associer à la définition des outils et des critères les principaux intéressés-

que ce dispositif représente pour l'avenir du logement social tel que nous le concevons, c'est-à-dire à vocation non résiduelle. Plus qu'un débat technique, il s'agit ici de dénoncer l'assèchement global et l'externalisation du financement des politiques publiques du logement, qui ont fait les frais depuis le début de ce quinquennat de la politique du rabot. Incarnée par la baisse des APL dès l'été 2017, cette politique s'est poursuivie avec la loi ÉLAN, marquant une étape supplémentaire vers la dérégulation, la marchandisation de ce secteur et la banalisation des acteurs du monde HLM, pourtant pivots des politiques publiques du logement. Cette loi a ainsi participé à soumettre le logement social à des logiques purement comptables, encourageant notamment la vente du parc HLM. Elle s'articule avec la réduction de loyer de solidarité engagée dans la loi de finances

Les lois de finances successives ont accompagné ce mouvement d'économies, estimées initialement à 1,5 milliard d'euros, puis ramenées à 800 millions les premières années et à 1,3 milliard sur la période 2020-2022.

Le référé de la Cour des comptes de décembre dernier a confirmé nos craintes, la Cour reconnaissant l'extrême fragilité dans laquelle ont été placés les organismes et bailleurs sociaux. Elle reconnaît le caractère injuste de ce mécanisme, puisque sa charge a davantage affecté les offices publics HLM, qui accueillent une plus grande proportion de ménages modestes et qui pratiquent des loyers faibles.

nous sommes dubitatifs sur la capacité des bailleurs sociaux à participer, dans ces conditions, à la lutte contre la précarité énergétique. Un ménage sur cinq est pourtant en situation de précarité énergétique dans notre pays ! Par ailleurs,

Face à ce constat implacable, nous estimons que les réponses formulées sont décevantes et ne constituent nullement des pistes sérieuses d'évolution. Pourtant, l'urgence est là et les chiffres sont parlants. Il n'y a jamais eu aussi peu d'agréments de logements sociaux : seuls 87 500 logements sociaux ont été agréés en 2020, soit une baisse de 17 % par rapport à 2019. En parallèle, le mal-logement touche désormais 4 millions de nos concitoyens. Pour remédier à cette situation, un nouveau protocole d'engagement a été signé le 19 mars dernier entre l'État et les bailleurs HLM : il fixe les objectifs de construction à 250 000 logements en 2021 et 2022. Pour rendre crédible cet engagement, nous pensons qu'il faut changer de braquet et donner concrètement aux organismes sociaux les moyens de remplir leur mission d'intérêt général au service du droit au logement pour tous, un objectif à valeur constitutionnelle. À nos yeux, ce changement de paradigme passe par un retour pérenne de l'État dans le financement des aides à la personne, mais aussi dans celui des aides à la pierre, qu'il a totalement abandonnées. Il faut cesser de ponctionner le 1 % Logement pour compenser ces désengagements. Par ailleurs, le secteur du logement fonctionne depuis un siècle sur deux jambes une publique et une privée. Cet équilibre doit être maintenu et les organismes HLM soutenus dans leur diversité. D'autres leviers doivent pouvoir être utilisés : réduction de la charge foncière, mais également révision de la loi SRU afin de la renforcer. Dans ce cadre, et alors que les objectifs de mixité sont plus que jamais d'actualité, nous regrettons que le projet de loi 4D prévoie de reporter à 2031 les objectifs de construction. Le séparatisme se situe aussi à ce niveau-là Pour conclure, mes chers collègues, nous espérons que le Gouvernement entendra la demande, quasi unanime sur les travées du Sénat, d'abandonner la RLS, à l'heure où nous avons plus que jamais besoin de politiques sociales et écologiques dans lesquelles le logement prend une place essentielle. D'autres pays, comme

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, s'il y a bien une réforme qui fait toujours autant débat depuis sa mise en oeuvre il y a trois ans, c'est bien celle Nous pouvons nous satisfaire de la finalité de cette réforme, qui visait à réduire les loyers des foyers occupant un logement social et percevant de trop faibles revenus. Mais derrière cette intention plus que louable se cachent des mécanismes financiers et opérationnels que nous

qui la supportent, en se faisant ponctionner en net : cela représente aujourd'hui près d'un milliard d'euros, soit en moyenne 5 % des loyers. Force est de constater que ce dispositif revient à faire financer par les bailleurs sociaux une diminution de l'engagement de l'État dans les APL.

Pour l'office départemental, Partenord Habitat, la réforme se traduit par une perte annuelle de 10 millions d'euros de fonds propres en loyers ponctionnés au titre de la RLS, pour un parc de 47 000 logements. Cela

pour l'habitat (ESH) de près de 30 000 logements, la réforme s'est traduite par une perte nette de 18,4 millions d'euros depuis 2018, l'équivalent de 440 logements neufs qui auraient pu être construits et qui ne l'ont pas été

ces collectivités. Nombre d'entre elles ont anticipé ce risque, en octroyant dans le cadre de conventions pluriannuelles un soutien financier substantiel. J'en veux pour preuve le soutien de la Métropole européenne de Lille à son office, LMH : il s'élève à 114,4 millions d'euros sur une période de dix ans, notamment pour faire face à la mise Il est aussi une évidence que nous ne pouvons pas nier : l'impact de la RLS sur les capacités d'investissement des bailleurs sociaux et l'effort consenti par les collectivités de rattachement des offices publics

les partenaires sociaux et Action Logement sont au rendez-vous. Ne pourrions-nous pas concevoir un État aux côtés des bailleurs sociaux pour relever ce défi, en repensant et en ajustant la RLS dans certains territoires ? Le second défi est la construction de 250 000 logements sociaux en deux ans. Le protocole d'engagement signé le 19 mars

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si nous sommes appelés aujourd'hui à débattre de l'effet de la réduction de loyer de solidarité mise en place par la loi de finances pour 2018, c'est bien que cette réforme pose problème. Un rappel au préalable : la RLS visait à réduire le coût des APL pour l'État.

Trois ans plus tard, quel bilan peut-on tirer de cette réforme ? Si l'on se fie au rapport de la Cour des comptes sur le sujet, il n'est guère brillant ! On relève trois défaillances une fragilisation des bailleurs sociaux et de leurs actions, tant en matière de construction que de réhabilitation du parc existant ; une mise en oeuvre qui, si elle a été progressive, n'en a pas moins soulevé d'importantes difficultés ; au bout du compte, des économies moins importantes que prévu pour l'État en raison de dépenses supplémentaires pour soutenir les bailleurs. Bien que nous manquions encore de recul pour évaluer à ce stade tous les effets de la RLS, la clause de revoyure prévue pour 2022 oblige à préparer ce réexamen dès à présent, en cherchant un point d'équilibre entre les besoins des bailleurs sociaux, l'objectif d'économies budgétaires pour l'État et la nécessaire simplification du dispositif. Rappeler aujourd'hui quelques-unes des erreurs stratégiques qui ont présidé à la mise en place de cette politique publique peut nous permettre, je l'espère, d'éviter qu'elles ne se reproduisent. C'est d'abord l'absence de concertation préalable avec les bailleurs sociaux qui a rendu la situation très difficile. Au-delà des débats parlementaires très vifs que nous avons pu avoir, notamment au Sénat, lors de l'examen du projet de loi de finances a obligé l'État à mettre en place des mesures d'accompagnement qui ont amputé l'économie budgétaire initialement prévue. Faute d'une négociation en bonne et due forme avec les organismes de logement social, la soutenabilité financière des conséquences pour eux de ce dispositif n'a pas été correctement analysée.

Enfin, cette réforme complexe a été difficile à mettre en oeuvre, le temps que les organismes sociaux se dotent des outils informatiques adéquats. tenu de cette impréparation initiale, les bailleurs sociaux craignent, à raison, que ce schéma de fonctionnement ne se reproduise l'année prochaine, après la clause de revoyure, et que leur situation ne s'aggrave davantage. En prévision de la négociation qui s'ouvrira en 2022, on ne peut que préconiser un dialogue avec l'ensemble des acteurs du logement social très en amont de l'échéance.

Même si la RLS n'est pas l'unique frein, il serait tout à fait malvenu de bloquer davantage les marges de manoeuvre des bailleurs et de réduire encore leurs capacités de construction et de rénovation. À cet égard, les objectifs d'engagements réciproques, qui, pour la période 2020-2022, montant des économies à réaliser grâce à la RLS ne devront pas suivre la même trajectoire exponentielle. Nous ne pouvons donc qu'encourager le Gouvernement à engager le plus rapidement possible une concertation réfléchie et constructive avec les organismes du logement social dans leur ensemble pour revenir sur cette réforme peu lisible, coûteuse dans sa gestion, et qui pénalise la construction de logements. Dans un premier temps, il importe de revenir sur la baisse des APL pour tenir compte du contexte économique actuel et des difficultés accrues des Français. La parole est à M. Philippe Dallier.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, que dire de plus ? Qu'ajouter à tout ce que mes collègues ont dit, y compris Patricia Schillinger, certainement plus inquiète qu'elle ne l'a dit des effets de la RLS sur l'avenir et l'activité des bailleurs sociaux ?

ces mesures devaient être accompagnées, ce que personne n'a rappelé, de la vente d'au moins 20 000 logements sociaux par an. L'objectif n'a pas été atteint- on en est à la moitié -et il ne le sera probablement pas dans les années à venir. Quant à l'impact des économies d'échelle attendues du regroupement des bailleurs, nous n'en mesurons pas encore aujourd'hui les effets. Quels seront-ils à échéance de deux ans ou trois ans ? Nous verrons La Cour des comptes, dans le référé qu'elle a rendu fin 2020, évoque tous ces points. Elle souligne également l'impréparation qui avait prévalu lors de la mise en oeuvre de cette réforme et qui a certainement concouru au ralentissement de la construction en 2018 et en 2019. Madame le ministre, dans ce secteur, comme dans tous les secteurs de l'économie,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

réduire le coût pour l'État des aides personnelles au logement. Il s'agissait de diminuer le loyer de certains logements sociaux en contrepartie d'une diminution des APL. devait permettre à l'État d'économiser 1,5 milliard d'euros par an. Neutre pour les locataires, cette réforme devait être absorbée par les 254 offices publics de l'habitat. À titre de compensation, le taux du livret A était gelé pendant deux ans et les bailleurs pouvaient notamment bénéficier d'un étalement de leur dette auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que de prêts de haut de bilan. Repoussons la dette, ne la gérons pas ! Avec mes collègues du groupe Les Républicains, nous avions dénoncé une réforme pensée à Paris, sans concertation préalable avec les bailleurs sociaux ni analyse suffisante de ses conséquences sur la construction de logements sociaux.

le gel des loyers en 2018 ou encore l'augmentation du taux de TVA de 5,5 % à 10 % sur la plupart des opérations de construction de logements sociaux. Dès octobre 2018, le président de l'Union sociale pour l'habitat (USH) tirait la sonnette d'alarme, dénonçant l'effondrement de la programmation des logements sociaux et de l'accession sociale. Revu à la baisse, le rendement des économies réalisées sur les APL grâce à la RLS a finalement été limité à 800 millions d'euros par an pour 2018 et 2019,

Le 4 mars dernier, la Cour des comptes a rendu public un référé qui, sans surprise, pointe les difficultés de mise en oeuvre de cette réforme,

financiers pour les bailleurs sociaux. Si le dispositif devait être neutre pour les locataires, en pratique, il ne l'est pas. À la fin de 40 000 foyers avaient déjà bénéficié d'une réduction de loyer sans être allocataires des APL. Or, qui dit bénéficiaires du système, dit nécessairement rupture d'égalité entre locataires. Selon la Cour, les bailleurs sociaux ont été privés de 4,5 % du montant des loyers. Si, dans un premier temps, ces derniers ont pu amortir cette baisse de ressources, les signaux d'alerte se multiplient réduction des investissements, ralentissement dans la production de logements neufs, retards dans la réalisation des engagements du programme de rénovation urbaine. En 2020, seuls 90 000 logements ont été construits sur les 120 000 qui

Une récente étude de l'OCDE montre que la part des revenus consacrée au logement est en augmentation depuis plusieurs années et qu'elle atteint en moyenne 37 % du budget des ménages très modestes. Développer une offre de logements abordables est ainsi essentiel à la vie de la Nation. C'est ma priorité en tant que ministre du logement et c'est la raison d'être du logement social. Nous le savons, plus de 70 % des Français sont éligibles au logement social et près de 2 millions de ménages sont encore en attente d'y accéder. Il est donc essentiel que les bailleurs sociaux mobilisent leurs moyens pour investir dans la construction et dans la rénovation. Alors que Alors que la Nation consacre plus de 5 milliards d'euros par an au logement social, l'État a mené plusieurs réformes structurelles visant à concilier soutenabilité de la dépense publique et ambition en matière de développement de l'offre de logements. La loi ÉLAN prévoit ainsi une profonde réorganisation en imposant aux organismes de gérer ou d'appartenir à un groupe gérant en cumulé au moins 12 000 logements sociaux. Cette mesure a pour principal objectif d'accroître et de dégager des marges de manoeuvre financières en réalisant des économies d'échelle et en optimisant l'utilisation des ressources du secteur et des organismes. Elle a également pour objectif de renforcer la professionnalisation des organismes, notamment sur les missions de maîtrise d'ouvrage ou d'ingénierie financière. Je suis avec attention ces regroupements. À ce stade, les trois quarts des organismes respectent cette obligation ou sont en voie de finaliser leur projet de regroupement.

de sa mise en oeuvre, laquelle a fait l'objet d'une large concertation avec les bailleurs et d'aménagements substantiels progressifs. La montée en charge du dispositif a notamment été étalée dans le temps : 800 millions d'euros en 2018, contre 1,5 milliard d'euros initialement prévus. un mécanisme de lissage entre les bailleurs a été mis en place par la Caisse de garantie du logement locatif social, afin d'assurer une juste répartition de l'effort entre les organismes. Il s'agissait, en particulier, de faire en sorte que les organismes qui logent les populations les plus précaires ne soient pas les plus touchés par cette réduction de loyer. Par ailleurs, des mesures d'accompagnement massives ont été mises en place par l'État,

À cela se sont ajoutés le gel du taux du livret A puis la révision de sa formule de calcul. Ces mesures bénéficient équitablement à l'ensemble des organismes de logement social, pour un gain annuel de 1,2 milliard d'euros en 2019. Les travaux de la clause de revoyure en 2019 entre l'État, les bailleurs, Action Logement et la Caisse des dépôts et consignations ont d'ailleurs montré que toutes ces mesures avaient permis de compenser intégralement l'effet de la RLS et de la TVA sur le compte de résultat des organismes J'entends les inquiétudes que vous avez tous exprimées, sur toutes les travées de cet hémicycle, sur les conséquences qu'aurait pu avoir la RLS sur la capacité d'investissement des bailleurs sociaux et donc sur la production et la rénovation de logements sociaux. Pourtant, en 2018 et 2019, soit les premières années de mise en oeuvre de la RLS, l'activité du secteur HLM s'est maintenue, les niveaux d'agrément ayant été assez élevés, entre 105 000 et 110 000 par an, en particulier pour les PLAI.

Vous conviendrez avec moi que l'on ne peut pas mettre les résultats de 2020, qui sont effectivement très décevants, sur le compte de la RLS. Ces résultats sont d'abord liés à la crise sanitaire et au délai de renouvellement des exécutifs municipaux, qui ont ralenti le dépôt des dossiers et leur instruction. Nous avons d'ailleurs eu le même problème avec les permis de construire en général et les mises en chantier de l'ensemble des logements, ce qui n'est pas imputable à la RLS. de contrôle du logement social (Ancols), publié le 25 novembre dernier, et l'édition 2020 de l'étude sur le logement social de la Banque des territoires, publiée en septembre 2020, ont par ailleurs montré que la situation financière des organismes HLM est bonne, même après la mise en oeuvre de la RLS, et que ce secteur dispose toujours d'une forte capacité d'investissement. Plus précisément, ces analyses ont montré que la capacité d'autofinancement par rapport au chiffre d'affaires est restée stable, de même que le ratio de ressources internes par rapport à la dette. Les ressources du secteur progressent en fait plus vite que l'endettement et le fonds de roulement net global reste élevé. Il est également à noter que les coûts de gestion par logement ont diminué en 2018 et 2019, après plusieurs années de hausse. Cependant, comme la Cour des comptes l'a souligné dans un récent référé, qui a été abondamment évoqué, il est vrai que les effets de la RLS ne peuvent encore être pleinement mesurés. Mon ministère s'attache donc à en suivre les conséquences, que ce soit sur la situation financière du secteur du logement social, sur la politique d'investissement ou sur les organismes les plus fragiles. Une nouvelle clause de revoyure est prévue afin d'étudier d'éventuelles modifications de ce dispositif. Comme cela a été indiqué à la Cour, je suis toute prête à étudier rapidement, d'ici à la fin de l'année, tout ce qui permettra de diminuer les irritants et les frais de gestion du dispositif pour les bailleurs, notamment s'il s'agit de limiter l'application du dispositif aux seuls allocataires des Au-delà de la clause de revoyure prévue concernant la RLS, le Gouvernement mène une politique ambitieuse de développement de l'offre de logement social pour les années qui viennent. Il faut déjà à tout prix rattraper l'année 2020. À cet égard, j'ai souhaité faire de 2021 et 2022 des années de mobilisation générale pour le logement social. C'est tout le sens du protocole en faveur de la relance de la production de logements sociaux que nous avons signé au mois de mars avec l'Union sociale pour l'habitat (USH), la plupart des fédérations HLM, Action Logement et la Banque des territoires. Ce protocole porte effectivement des objectifs très ambitieux : l'agrément de 250 000 logements sociaux sur deux ans, en 2021 et 2022, dont 90 000 logements très sociaux. Des moyens exceptionnels seront mobilisés par l'État, par Action Logement, par la Caisse des dépôts et consignations sur la même période. Cela passe par un soutien de l'État de 500 millions d'euros à la réhabilitation lourde des logements sociaux dans le cadre du plan de relance, une mobilisation accrue du Fonds national des aides à la pierre, mais également par une hausse de 920 millions d'euros des financements du secteur par Action Logement, dans le cadre de l'avenant à la convention quinquennale signé le 15 février dernier, et par la distribution de 200 millions d'euros de titres participatifs supplémentaires de la Caisse des dépôts et consignations, portant le total à 1 milliard d'euros, pour renforcer les fonds propres des organismes. J'ai tenu à mettre en place une gouvernance renforcée de la mise en oeuvre de ce protocole afin d'assurer le suivi des engagements de chacun et la déclinaison opérationnelle dans les territoires.

Nous avons fait le choix d'inscrire des dispositions en ce sens dans le projet de loi 4D, afin d'assurer la pérennité du dispositif SRU au-delà de 2025, tout en l'adaptant aux réalités territoriales. Grâce aux propositions de la commission nationale SRU et à une concertation avec les associations de collectivités locales, je pense que nous avons atteint un dispositif équilibré, lequel sera très bientôt soumis à votre examen. Agir pour le logement social passe également par le déploiement d'une politique ambitieuse en matière de mixité, car c'est la clé de la cohésion sociale. Le projet de loi 4D portera des mesures en ce sens, notamment pour renforcer le rôle des EPCI en matière d'attribution et pour aider au logement des travailleurs clés. Ce projet de loi, enfin, permettra de reporter, au plus tard à la fin de 2023, la mise en oeuvre de la cotation de la demande et de la gestion en flux, compte tenu des difficultés liées notamment à la crise du covid-19 et au renouvellement des exécutifs locaux. En conclusion, mesdames, messieurs les sénateurs, je dirai que le logement social a été au rendez-vous de la crise que nous traversons, qu'il a joué son rôle d'amortisseur social et qu'il s'est adapté afin de mieux accompagner ses locataires. Le logement social est un facteur clé de la cohésion du pays ; le mouvement HLM est un partenaire essentiel pour l'État. Le Gouvernement fait de l'avenir de ce secteur l'une de ses priorités. C'est pourquoi nous relançons la construction ; c'est pourquoi nous pérennisons la loi SRU, afin de permettre à chacun d'avoir accès à un logement abordable.